Le Gouvernement revient aujourd'hui devant nous pour la troisième fois en trois semaines avec des propositions de modification en profondeur de son projet de budget pour 2019. Dont acte, compte tenu de la situation sociale dans le pays. Nous voterons d'ailleurs une grande partie des nouvelles mesures. Mais je veux relever que cette désorganisation des travaux budgétaires aurait pu être évitée si le Gouvernement avait tenu compte plus tôt des propositions exprimées, ici ou ailleurs, par les différents groupes parlementaires qui composent la Haute Assemblée. À nos À nos propositions, qui ont pu concerner la prime d'activité, la CSG des retraités et bien d'autres mesures, le Gouvernement nous a systématiquement et seulement répondu : « Halte aux dépenses !

Je veux donc dire au Gouvernement qu'à l'avenir, lors des prochaines discussions budgétaires, et en premier lieu pour les budgets rectificatifs, qu'on annonce nombreux, il serait bienvenu d'écouter, d'entendre les parlementaires et leurs propositions et d'entrer pleinement dans le débat. C'est en nous respectant, monsieur le ministre, que vous réussirez à écrire une bonne loi, et notamment celle du budget, pour notre pays, la France. Écoutez, entendez, quand des alternatives vous sont proposées, et vous éviterez peut-être ces contradictions si nombreuses entendues au banc des ministres depuis trois semaines au rythme des annonces faites depuis l'Élysée

laisser penser qu'il a entendu la colère populaire, céder le moins possible et, surtout, jusqu'au bout, ne faire participer ni les riches ni les entreprises au moindre effort national. Il a annoncé mot pour mot une « augmentation du SMIC de 100 euros », sans préciser qu'il s'agissait de 100 euros bruts et que

Tout montre que ce seront les contribuables, y compris les plus modestes, qui devront mettre la main à la poche, alors que les riches et les ultra-riches seront toujours protégés. Ce n'est pas d'une part, il n'y a pas d'augmentation de salaire- seuls 2 à 3 millions de salariés seront concernés par l'anticipation que j'évoquais -et, d'autre part, toutes les nouvelles dépenses seront prises en charge par la collectivité. Emmanuel Macron, passant du tour de passe-passe au numéro d'équilibriste, a tenté d'expliquer l'inexplicable : le refus de rétablir l'ISF pour les financiers et actionnaires de tout poil. l'ISF est, pour les « gilets jaunes » et pour la grande majorité de la population qui les soutient, le marqueur d'une politique dont la priorité est la satisfaction non pas des intérêts du plus grand nombre, mais de quelques intérêts privés. privés. Nous le disons avec force au chef de l'État mais aussi à la majorité sénatoriale : rendez l'ISF ! Rendez ces 3,7 milliards d'euros pour participer à la justice fiscale et sociale Rendez l'ISF, pour apporter un moindre crédit à cette idée de « nouveau contrat social », qui sonne aujourd'hui comme un simple affichage de la part d'un pouvoir s'appliquant, par ailleurs, à poursuivre avec zèle la déconstruction du modèle social. donc à demander une seconde délibération sur l'article 82 du projet de loi de finances, relatif à la prime d'activité. Monsieur le président, notre groupe estime que, pour la clarté des débats et des choix, une seconde délibération sur les dispositions relatives à l'impôt sur la fortune devrait avoir lieu. Notre peuple a le droit de savoir en effet qui va payer les dispositions annoncées hier par Emmanuel Macron

il y a cette idée que la France, championne d'Europe de la dépense fiscale, crée toujours plus de taxes et d'impôts qui grèvent finalement le pouvoir d'achat des Français. Il y aura moins d'impôts et moins de taxes lorsqu'il y aura moins de dépenses publiques, c'est une évidence

j'ose dire, à une crise des conditions matérielles. Elle est aussi un cri existentiel : les Français pensent qu'ils ne comptent plus et que, comme le disait Jacques Julliard, la démocratie se fait sans le peuple.

de Françaises et Français qui manifestaient, qui apportaient leur soutien aux manifestations ou qui s'interrogeaient simplement sur le devenir du pays, le Président de la République a fait hier un certain nombre d'annonces très importantes,

Par ailleurs, le Gouvernement a bien une ligne de conduite qu'il va suivre une nouvelle fois, y compris dans la discussion parlementaire : il ne pourra pas y avoir, car nous ferons attention à nos comptes publics, de dépenses publiques supplémentaires. Si le déficit public se creuse par l'effet des mesures, notamment de baisse de fiscalité, annoncées par le Président de la République, chacun constatera qu'il ne s'agira pas de dépenses publiques supplémentaires. Le Président de la République hier n'a pas proposé de dépenses publiques supplémentaires

Que se passe-t-il du côté des comptes publics ? Le Gouvernement a proposé au Parlement, au début de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances de l'État et des collectivités locales, un déficit public, toutes administrations publiques confondues, de 1,9 %.

Mais le déficit public présenté dans nos documents budgétaires au Haut Conseil des finances publiques, au Parlement et à la Commission est de 1,9 %. À la fin des débats parlementaires, au moment même où le Président de la République prenait la parole, le Parlement, et- permettez-moi de le souligner -principalement le Sénat, a dégradé la copie des comptes publics de 0,1 point, c'est-à-dire à peu près 2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires- soit autant de recettes en moins,

Nous sommes bien d'accord qu'il ne s'agit pas de recettes sur lesquelles le Gouvernement s'assoit, puisque cette prime n'existait pas et n'était pas défiscalisée. On peut penser qu'il y a, en revanche, ici ou là, quelques effets d'aubaine qu'il nous faudra chiffrer, mais qui ne sont pas de nature à bouleverser l'équilibre des comptes publics. Donc, du du côté des comptes publics et de la présentation du débat budgétaire, puisque le président Kanner nous a appelés à la sincérité des documents et des débats, nous en sommes aujourd'hui, avec l'annonce du Premier ministre de l'arrêt de la taxation carbone et les annonces du Président de la République, à 10 milliards d'euros, soit 0,5 point de dégradation des finances publiques.

il s'agit d'une accélération de trajectoire, mais il n'y a pas d'augmentation de la dépense publique. C'est une baisse de la fiscalité qui explique, en effet, la dégradation des comptes publics et le 2,5 % de déficit, alors que le Gouvernement vous a proposé une copie à 1,9 % lorsqu'il vous a présenté ses documents budgétaires.

Dès l'année dernière, le Sénat avait gelé les tarifs de TICPE au niveau de 2017. Cette année, nous avons introduit un article additionnel visant à maintenir les tarifs au niveau de 2018. D'ailleurs, le Gouvernement devrait

semble-t-il, à l'unanimité du Sénat, notamment sur l'arbitrage de dividendes, que vous n'avez pas voulu chiffrer. Nous avons également eu un désaccord sur le coût des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties à la charge des collectivités.

Pour ces raisons de désaccord profond sur les chiffrages, nous avons été amenés à refuser l'article d'équilibre. Nous avons voté l'ensemble des articles de la seconde partie, en finissant hier soir, et dans

Je rappelle au Sénat les termes de l'article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission,

d'exposer aujourd'hui, dans l'une des assemblées, sans doute à l'Assemblée nationale, les mesures de façon pédagogique. Pour l'instant, cela n'a pas été fait. Monsieur le ministre, je pense que vous devez au peuple français une explication claire et nette sur le contenu de ces mesures

Nous ne pouvons qu'être favorables à une revalorisation de la prime d'activité. C'est d'ailleurs une mesure que nous avons proposée très récemment, dans la proposition de loi visant à répondre à la colère des pour plus de justice et d'égalité, déposée le 3 décembre dernier par les députés et les sénateurs socialistes afin de sortir de la crise. Nous pensons que cette mesure est utile et doit être accompagnée d'une réflexion sur le réalignement vers le haut des salaires supérieurs au SMIC.

Enfin, la question du financement doit être posée, car elle a été complètement occultée à ce stade. La modification de l'article que nous voterons ne doit pas avoir pour conséquence la mise en place d'un mécanisme de bonneteau fiscal, qui aboutirait à reprendre d'une main ce qui est donné de l'autre.

La colère de ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois est tout à fait légitime. À quoi correspond ce geste ? Il semble, d'après ce que nous comprenons, que les 100 euros de hausse du SMIC net correspondent à une revalorisation couplée à une baisse des charges de 30 euros. Monsieur le ministre, je ne sais pas si la formule que vous nous proposez est la bonne. Ce qui est certain, c'est qu'elle semble la moins mauvaise. Pourquoi ?

Nous voterons la hausse. Comment nous y opposer ? Toutefois, nous souhaitons que ses effets soient évalués et fassent, le cas échéant, l'objet d'un lissage, pour que les personnes touchant plus que 1,2 ou 1,3 SMIC ne soient pas lésées.

Naturellement, je veux le dire à mon tour avec l'esprit de responsabilité qui caractérise les membres de cette assemblée, notre groupe votera consécutivement les amendements et le budget, mais chacun d'entre nous sait très bien qu'il va falloir revenir sur ces lignes, somme toute assez confuses.

d'activité est calculée, on le sait, au regard des deux salaires dans la famille, compte tenu des allocations logement et de toute une série d'aides. Ce n'est pas une rémunération du travail, c'est une aide publique pour compenser l'insuffisance des salaires. Je ne crois pas que les Français attendent aujourd'hui qu'une aide publique payée en vidant les caisses de la sécurité sociale se substitue à une nécessaire revalorisation de leur salaire. Cette prime d'activité, il faut la demander

Le scrutin est clos.

Avant de passer au vote sur l'ensemble du texte, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits par les groupes pour expliquer leur vote. J'indique au Sénat

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour mettre un peu d'humour dans une actualité dans une actualité qui ne porte pas à sourire, souvenez-vous de cette déclaration fiscale présentée sous forme musicale : « On est là pour te pomper, « T'imposer sans répit et sans repos. « Pour te sucer ton flouze, « Ton oseille, ton pognon, « Ton pèze, ton fric, « Ton blé, tes économies, tes sous, « Ton salaire, tes bénéfs, « Tes bas de laine, « Tout c'qui traîne.

cette chanson, cette réalité d'hyper-fiscalité, ne fait plus rire personne. Avec 9 millions de pauvres, des centaines de milliers de nos compatriotes dans la rue depuis des semaines, vêtus de leur gilet de détresse, l'heure est grave pour notre pays. Elle l'est d'autant plus que le Président de la République a confirmé hier soir, dans son allocution solennelle, qu'il ne remettait pas en cause son système ultralibéral ni la mondialisation sauvage qui fabriquent chaque jour davantage de pauvres et toujours plus d'exclus. Alors que l'urgence est de répondre à la souffrance de millions de nos compatriotes, je voudrais souligner combien une mesure de ce projet de loi de finances version « Haute Assemblée » montre qu'Emmanuel Macron peut compter sur l'appui de la majorité sénatoriale pour servir les intérêts de quelques-uns, de quelques amis influents, au détriment du plus grand nombre. Pendant que les « gilets jaunes » battaient le pavé, le Sénat et sa majorité, à savoir le groupe Les Républicains, ont en effet introduit des modifications dans ce PLF pour exonérer d'impôts non pas les classes moyennes, ni même les smicards, mais les grands médias. Ce sont 50 millions d'euros qui ne rentreront plus dans les caisses de l'État ; ce sont 50 millions d'euros volés dans la poche des Français ! Cette exonération de taxes pour les grands médias audiovisuels était-elle à ce point urgente et si justifiée ? Elle confirme néanmoins que vos grandes déclarations ne sont que des postures et nous rappelle que, lorsque la droite était au pouvoir, rien n'a été fait pour baisser la dépense publique, rien n'a été fait pour retrouver notre souveraineté budgétaire ni pour baisser la fiscalité. Chez Les Républicains, à l'image de M. Wauquiez et de son gilet jaune, on est frappé d'amnésie sélective. Au lieu d'insuffler l'espoir en l'avenir et de laisser entrevoir un horizon d'optimisme français, tous les partis politiques ont préféré faire de 2019 l'année du racket fiscal et du « pire qu'avant Preuve en est, hier, une heure avant l'intervention du chef de l'État, le vote du Sénat sur l'allégement de l'qui sanctionnait les exilés fiscaux.

Vous en conviendrez, monsieur le ministre, ce débat s'est déroulé dans un drôle de contexte : un climat de révolte comme nous n'en avions plus connu depuis mai 68. Votre budget initial, comme celui de l'an dernier, était le reflet d'une politique qui n'est aujourd'hui pas comprise par une grande majorité de nos compatriotes, celle qui s'exprime bruyamment et parfois- malheureusement -violemment. Elle n'est pas comprise non plus par ceux qui s'expriment moins, mais qui doivent avoir toute notre attention les chômeurs et les plus pauvres. Les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat. Nous avons, et depuis longtemps, des problèmes budgétaires. Ces deux séries de problèmes sont liées.

Ce contexte, c'est aussi un mutisme quasi total de Bercy en matière de chiffrage de nos propositions. En nous obligeant, la plupart du temps, à amender au doigt mouillé, le Gouvernement s'offre des arguments faciles pour s'opposer à nos suggestions. Ce fut notamment le cas lorsque nous avons proposé de réformer en profondeur l'impôt sur le revenu ou encore les droits de succession. À défaut d'informations, nos marges de manoeuvre sont très limitées. Pourtant, si nous manquons d'informations et de moyens, notre sens de l'initiative, lui, ne manque pas de ressources. Le Gouvernement aurait été bien avisé de s'inspirer des travaux de tous nos collègues. Le travail réalisé ici est de qualité. Utilisez-le, monsieur le ministre Nous avons ainsi réussi à améliorer sensiblement ce budget, malgré votre opposition quasi systématique. Laissez-moi vous donner quelques exemples : suppression des petites taxes : avis défavorable du Gouvernement relèvement du quotient familial : avis défavorable ; simplification de l'impôt sur les plus-values immobilières : avis défavorable ; facilitation de la transmission d'entreprises : avis défavorable ; économies sur le temps de travail et les jours de carence dans la fonction publique : avis défavorable gel de la fiscalité sur les carburants : avis défavorable, avant que vous ne finissiez- bien tard, malheureusement -par revenir dessus ; lutte contre l'arbitrage des dividendes : enfin un avis de sagesse, mais il est vrai que cette mesure peut rapporter entre 1 milliard et 3 milliards d'euros. Nous avons décidé très tôt, ici, au Sénat, de supprimer la hausse des taxes sur les carburants. À un moment où le Gouvernement s'entêtait encore, malgré la colère des Français. Si nous l'avons fait, c'est parce que notre expérience d'élus locaux et notre connaissance du terrain nous ont convaincus que les Français n'en peuvent plus du toujours plus d'impôts. Ce que nous apprend notre expérience d'élus locaux, nous qui avons vécu et géré des revendications et des conflits, c'est qu'un incendie, ça s'éteint dès le début et le plus rapidement possible. L'expérience, monsieur le Après les annonces du Président de la République, on pourrait considérer que votre budget est devenu,, insincère et ne pas le voter. Toutefois, le groupe Union Centriste entend saluer le sens de l'anticipation et la sagesse du Sénat. Nous voterons donc pour ce budget largement amélioré par notre assemblée. J'ai abordé le contexte et le contenu, voyons maintenant les perspectives. Que faut-il faire aujourd'hui ? Votre budget ne prévoit ni baisse des dépenses ni refonte globale de notre fiscalité. Or, s'il est une leçon que nous apprennent les quarante dernières années, c'est que plus de dépenses, c'est forcément plus d'impôts. C'est bien ce qui est inquiétant dans les annonces du Président de la République, qui viennent s'ajouter à celles du Premier ministre : 12 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, ce sont forcément 12 milliards d'euros d'impôts supplémentaires à court terme. Certes, il est quelque peu injuste d'hériter de quarante années de laxisme budgétaire.

Elle nécessite une démarche juste, équilibrée, courageuse, à laquelle nous sommes prêts. Depuis 2006, la dépense publique a augmenté de 300 milliards d'euros. Elle augmente beaucoup plus que la population et l'inflation cumulées. Pourtant, les Français ont le sentiment que le service public se dégrade. C'est un paradoxe très grave pour la démocratie : on dépense de plus en plus et les services publics sont perçus comme de moins en moins performants. Il est grand temps d'inventer le service public du XXI siècle : plus modeste, plus moderne, plus efficace et moins coûteux.

concerne les recettes, il est temps de s'attaquer au scandale des GAFA et d'autres entreprises qui paient très peu d'impôts, si ce n'est pas du tout. En la matière, la France doit reprendre la main si l'Europe continue de traîner autant les pieds. que dire du nécessaire renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et sociale ? C'est une question à laquelle nous sommes très attachés ici, au Sénat. En témoigne l'initiative du groupe Union Centriste contre les fausses inscriptions au répertoire de l'INSEE- 1,8 million de faux Nathalie Goulet. En tout cas, le Gouvernement n'a pas mis à profit l'embellie de la conjoncture pour assainir nos finances. Monsieur le ministre, l'heure est grave, mais il n'est pas encore trop tard si nous refusons de tomber dans la facilité en opposant les ruraux aux urbains, les retraités aux actifs, les héritiers aux non-héritiers, les collectivités à l'État. Nous devons, au contraire, faire le choix de la responsabilité et du courage, en déterminant collectivement les dépenses que nous sommes prêts à baisser, et en accepter les conséquences. Cette démarche ne pourra aboutir que si l'on y associe l'ensemble des Français, en particulier les corps intermédiaires, tant négligés depuis le début du quinquennat. Monsieur le ministre, vous avez devant vous des élus de bonne volonté, des élus de la République, des représentants du peuple, et non pas seulement des collectivités. Sur toutes les travées, dans notre diversité qui est celle du peuple français, notre travail est reconnu comme étant de qualité.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous terminons l'examen du deuxième projet de loi de finances du quinquennat dans un contexte difficile, qui tranche sensiblement avec la situation de l'année dernière. Le Président de la République s'est exprimé hier soir. Il a annoncé des mesures fortes en faveur des salariés et des retraités les plus modestes, qui rendent la poursuite des violences encore plus inacceptable. Ceux qui appellent à les prolonger sont non seulement irresponsables, mais aussi incohérents. Ils mentent aux Français. Comment expliquer « en même temps »

Où est la cohérence ? Mes chers collègues, il faut maintenant cesser la surenchère. Dans ce contexte de crise politique et sociale, le risque serait dorénavant de revoir nos ambitions à la baisse, de faire l'autruche, de faire comme nous avons toujours fait, à savoir augmenter les dépenses et les impôts. Au contraire, nous croyons que le temps des vieilles recettes est révolu et qu'il faut faire preuve de responsabilité. C'est valable pour les « gilets jaunes », pour les parlementaires et pour le Gouvernement.

Hier, le Président de la République a fait preuve de lucidité face au déclassement social d'une partie de nos concitoyens et à l'érosion continue de leur pouvoir d'achat depuis plus de vingt ans. Mais le mal est plus profond. C'est de l'essoufflement du « modèle français » qu'il est question. Ce modèle rime aujourd'hui avec un État obèse, des services publics de plus en plus éloignés et une hausse des inégalités. Pour répondre à cette détresse, le Sénat a fait plusieurs propositions lors de l'examen de ce budget, en direction des personnes modestes et des petites entreprises : gel de la hausse de la TICPE,

celle des élus locaux, des élus ruraux, qui se sentent trop souvent ignorés par l'État. Ils sont au plus près des citoyens, ils leur ont ouvert leurs portes ces derniers jours, comme à leur habitude, pour comprendre leurs inquiétudes. ces élus ne demandent qu'une chose : les moyens d'agir. Le Sénat, là encore, a sensiblement amélioré le texte du Gouvernement s'agissant des collectivités territoriales, pour mieux prendre en compte les spécificités locales. Il faut que le Gouvernement travaille avec les élus locaux dans les prochaines semaines : ils sont l'une des clés de la sortie de crise, car ils forment l'ossature de la République. L'autre responsabilité du Gouvernement, c'est d'engager l'indispensable refonte de la dépense publique et de la fiscalité de notre pays. Les annonces du Président de la République doivent maintenant être financées. Mais il serait insupportable et incompréhensible pour les Français que cela se fasse au prix de plus d'impôt et de plus de dette.

En punition, nous avons eu le pire des deux mondes : plus de dépenses publiques et moins de services publics ; plus de dette et moins de justice ; plus de mots et moins d'actes. Aujourd'hui, monsieur le ministre, il vous incombe de faire les réformes que tous les autres ont mises sous le tapis : repenser les mesures fiscales punitives et complexes héritées des quinquennats précédents évaluer - enfin ! -la dépense publique pour supprimer les programmes inefficaces ; réduire la dette et donner des perspectives d'avenir à nos concitoyens. Les événements nous mettent au pied du mur. Allons-nous sortir de cette crise, comme de tant d'autres auparavant, avec un rafistolage qui ne changera rien, ou bien profiterons-nous de cet électrochoc pour résoudre le mal français ? Nous l'avions dit lors de la discussion générale : ce budget est trop timide pour sortir la France de l'ornière. Il est d'ailleurs déjà caduc. Il est aujourd'hui de votre responsabilité, monsieur le Mais la responsabilité de la représentation nationale, particulièrement du Sénat, n'est pas moins grande, la dégradation du climat social étant propice à la démagogie, aux postures et au jusqu'au-boutisme. L'année dernière, en choisissant Emmanuel Macron plutôt que Marine Le Pen, les Français avaient envoyé à la classe politique un message de modération, d'apaisement des antagonismes et de préférence pour les propositions constructives. Cela n'était pas pour déplaire au Sénat, qui, sous l'égide de son président actuel, pratique largement ces vertus. Très bien ! C'était également la raison d'être de notre groupe. Aujourd'hui, alors que la crise gronde, souvenons-nous de cet appel. En temps de crise, la modération est un courage et un effort, dont nous montrer dignes. En ces temps difficiles, soyons force de proposition pour sortir notre pays de l'ornière dans laquelle il est bloqué depuis trente ans. Monsieur le ministre, nous voterons ce projet de loi de finances, à la condition qu'il soit la première étape d'une refondation plus large du modèle français. C'est une nécessité politique et sociale. Nous sommes prêts à participer aux concertations qui auront lieu dans les prochains mois pour réformer vraiment notre pays ! La parole

enfermés dans leurs certitudes et souvent perçus comme méprisants par nos concitoyens. L'année 2019 devait être celle du pouvoir d'achat. C'est l'heure de la preuve, la preuve que nous tenons nos promesses », disiez-vous, monsieur le ministre de l'action et des comptes publics, en septembre dernier. Quelle puissance de conviction !

l'augmentation des taxes sur les carburants, le gaz et l'électricité votée par vos prédécesseurs ? Rien de tout cela ne figurait dans le programme du Président de la République. Vous parliez Vous parliez pouvoir d'achat, mais vous repreniez d'une main ce que vous donniez de l'autre. Les grands perdants sont toujours les mêmes, à savoir les classes moyennes actives ou retraitées. Pour elles, depuis dix-huit mois, c'est un bonneteau fiscal dont elles n'ont pas été dupes. Cette fracture fiscale se double d'une fracture territoriale pour celles et ceux qui n'ont d'autres choix que d'utiliser leur voiture au quotidien. Cette fracture-là, vous n'avez pas non plus voulu Quant à l'ISF, autre sujet de controverse, vous l'avez partiellement supprimé, conservant cependant un impôt sur la fortune immobilière. Mais votre sans mesure de réorientation des capitaux, s'est traduite par une désertion des dispositifs qui finançaient nos PME, au profit, comme d'habitude, de l'assurance vie et des emprunts d'État. Vous avez ainsi perdu sur les deux tableaux celui de l'opinion, car l'ISF est un totem, et celui de la capitalisation de nos entreprises. Comment vous étonner que votre politique fiscale soit considérée comme injuste et inefficace par une grande majorité des Français ? ? En imaginant pouvoir confisquer, au profit du budget général de l'État, une grande partie des taxes dites « écologiques », vous avez de plus porté un coup à l'idée même de transition énergétique. La hausse des taxes sur les carburants a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la colère des Français. C'est leur consentement même à l'impôt, fondement de notre démocratie, que vous avez mis à mal. Tout cela en dix-huit mois : beau résultat Que n'avez-vous écouté le Sénat lorsque nous avons réindexé les retraites lors de l'examen du PLFSS ? Que n'avez-vous écouté le Sénat lorsque nous avons revalorisé le quotient familial et les prestations familiales ? Que n'avez-vous écouté le Sénat lorsque nous avons voté l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants ? tenté de vous alerter contre les effets calamiteux de votre politique du logement, qui est en train de plonger un secteur entier dans la crise ? Au lieu de cela, au moment du vote de la première partie de ce projet de loi de finances, vous avez fustigé l'irresponsabilité de la Haute Assemblée, accusée de creuser le déficit, avant même de voir quelles économies nous allions proposer.

Malgré tout, notre vote pour ce budget donnera à la majorité sénatoriale la satisfaction d'avoir montré la voie au Gouvernement sur bien des points.

tenir le déficit ou le laisser filer au-delà des 3 % du PIB, d'autant que la croissance risque manifestement de ne pas être au rendez-vous de vos attentes.

Faute d'avoir engagé, dès le début du quinquennat, les réformes structurelles nécessaires, il est malheureusement à craindre le retour du rabot budgétaire et le gel ou- pourquoi pas ? -le sur-gel des crédits votés. Quoi qu'il en soit, nous formons le voeu que ni le budget de nos forces armées ni celui de nos forces de sécurité ne figurent dans les variables d'ajustement budgétaire. Vous avez déjà, en PLFR, donné un coup de canif à la loi de programmation militaire. Nous devons maintenant sanctuariser ces deux budgets. C'est le minimum que nous devons aux hommes et aux femmes qui risquent leur vie pour défendre notre liberté, nos valeurs, notre République. Quant à la trajectoire 2018-2022, elle est morte hier soir. Elle n'intégrait déjà pas la suppression complète de la taxe d'habitation, qui coûtera 10 milliards d'euros de plus. Il faut maintenant financer les annonces du Président de la République. Dans un contexte de grande incertitude, où la remontée des taux d'intérêt devient chaque jour plus probable, nous ne pouvons pas abandonner l'objectif d'une inversion rapide de la courbe de la dette. Vous devez, monsieur le ministre, y apporter Le groupe Les Républicains votera ce projet de loi de finances modifié par le Sénat. Il rendra ainsi un grand service au Gouvernement, ne serait-ce que pour permettre à l'Assemblée nationale de maintenir l'annulation des taxes sur les carburants, de toucher à la prime d'activité et peut-être de confirmer d'autres mesures, notamment sur le

Nous sommes prêts, en responsabilité, à nous remettre au travail. Mais il est temps que vous changiez de cap. L'acte I du quinquennat est terminé. Le mirage du nouveau monde s'est dissipé. Le temps vous est compté, comme il est compté à la France

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous avons vécu, il est vrai, une séquence budgétaire assez inédite.

le contexte donne une coloration particulière à notre loi de finances. Une partie des modifications a déjà été prise en compte dans ce texte. Par honnêteté intellectuelle, je dois reconnaître une forme de clairvoyance à la majorité sénatoriale

pouvoir d'achat : les sujets sont sur la table. Le bicamérisme a joué son rôle et je sais que les territoires joueront leur rôle dans ce débat.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. vous avez la parole

soit 1 188 euros nets ; RSA, 550,93 euros pour une personne seule sans enfant et 1 157 euros pour un couple avec deux enfants ; minimum vieillesse, 634,66 euros pension de retraite moyenne des femmes, 1 091 euros bruts, inférieure de 42 % à celle des hommes. Voilà la réalité ! Voilà la vie réelle de millions de nos concitoyens, qui attendaient des réponses claires du chef de l'État à leur exigence de vivre mieux, d'être respectés dans leur dignité. Tout en maintenant son cap, le Président de la République, précédemment pour sa vision avant-gardiste de la politique, a rencontré l'humilité et reconnu, enfin, le légitime élan populaire citoyen qui souffle actuellement sur notre pays.

pour les plus petites retraites, pourtant refusé par le Gouvernement pendant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour le reste, rien qui n'effraiera les marchés financiers ou le grand patronat, exonéré de toute augmentation des salaires. Cela approfondira, soyez-en certains, la défiance populaire à l'égard des politiques gouvernementales. Qu'on en juge : pas de hausse du SMIC, gel du point d'indice des fonctionnaires, gel de l'allocation adulte handicapé jusqu'au 1avril 2020.

par la suppression de l'ISF, des évadés fiscaux protégés, des actionnaires libres de ponctionner les richesses produites par les salariés au détriment de leurs salaires. C'est ce que contient la loi de finances, reflet de la prise en compte, comme nous pouvons le voir, de la défense du pouvoir d'achat et de la juste rémunération du travail

Je ne reviens pas ici sur le fait que le Sénat a fini par arracher le gel des taxes sur les carburants, après avoir voté toutes les hausses antérieures. Le jeu de la commission mixte paritaire permettra au Gouvernement de revenir sur quelques mesures votées ici, donnant au texte final de la loi de finances sa pleine dimension ultralibérale. Les mesures annoncées hier dans l'allocution enregistrée du Président de la République ne changeront pas la donne, puisque la facture sera soldée par encore plus de droits indirects et de TVA et encore moins de services publics ! La politique du « fort avec les faibles, faible avec les forts », qui anime aujourd'hui un pouvoir désavoué,

Depuis le printemps 2017 et l'élection par défaut d'Emmanuel Macron et de sa majorité, si une forme de contrat a bien été passée, c'est directement avec la finance, avec les affairistes, pour mener une politique conforme à leurs intérêts égoïstes, bien loin de l'intérêt commun. Y figuraient en bonne place la réforme du code du travail par ordonnances, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'instauration de la sur les revenus du capital et du patrimoine, le nouvel allégement des droits de mutation et de succession, le démantèlement des services publics, de la SNCF et du secteur hospitalier,

Cette République du contrat avec la finance ne peut qu'engendrer des dommages collatéraux : chômage de masse, précarité du travail renforcée, tensions urbaines, désespoir rural, casse des services publics de proximité et stagnation des salaires. Pour que certains gagnent, il faut que d'autres perdent, et ce sont les plus nombreux. D'une colère très juste surgit une balbutiante espérance, jusqu'ici contrariée par les prétentions de la finance. L'Europe n'est pas capable d'agir comme il convient, en témoigne l'échec de la négociation sur la taxation des fameux GAFA. Nous ne savons pas mettre à contribution en France, puisqu'il suffit que la Fédération bancaire française fronce un sourcil pour que le Gouvernement s'exécute. Pourtant, avec des milliards d'euros de frais bancaires extorqués aux entreprises comme aux particuliers, avec les 2 600 milliards d'euros que la Banque centrale européenne a répandus ces dernières années

Il est temps de mettre de la démocratie dans cette société, où les droits sont mis en cause : démocratie dans les institutions, dans la cité, dans les entreprises, au sein de la sécurité sociale. démocratie partout ! C'est bien ce tournant démocratique qui surgit sous nos yeux, celui d'un peuple qui ne veut plus en rabattre sur ses aspirations au nom d'une prétendue « fin de l'Histoire avec le capitalisme financiarisé à outrance. Oui, tout le monde veut gouverner : les citoyens, les élus locaux, les parlementaires et même la jeunesse ! Et alors ? Enfin, je veux remercier tous les personnels du Sénat, sans exception, de leur précieux concours aux travaux de ce projet de loi de finances, que notre groupe va évidemment rejeter, sur le fond comme sur la forme. La

Notre pays se trouve dans une situation extrêmement troublée, marquée par un réel décrochage entre une grande partie de nos concitoyens et les acteurs de la vie publique, qu'ils soient syndicalistes, associatifs ou politiques, gouvernants comme opposants. Nous assistons à une contestation forte des politiques publiques par une large majorité de l'opinion publique, nourrie notamment par le sentiment d'accroissement des inégalités sociales, par le constat d'une iniquité fiscale qui s'accentue chaque année ou encore par l'aggravation des fractures territoriales. Le mouvement des « gilets jaunes » a bien d'autres facettes, mais reconnaissons que celles-là émergent clairement et doivent trouver un débouché dans nos travaux, au moment où nous examinons les textes financiers que sont le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances. En tant que parlementaires, représentants de la Nation, nous nous devons d'entendre cette révolte citoyenne et d'en nourrir nos réflexions et décisions. C'est dans cet esprit que les socialistes ont souhaité présenter un contre-budget ayant vocation à rediriger une partie des recettes vers le pouvoir d'achat des classes moyennes et de nos concitoyens les plus modestes. C'est encore dans cette optique que nous venons de déposer, la semaine dernière, une proposition de loi allant dans le même sens avec nos homologues de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, nous regrettons qu'il ait fallu attendre quatre semaines pour que le Gouvernement daigne vraiment s'intéresser à un mouvement populaire, certes protéiforme, mais représentatif de nombre d'angoisses et de colères aujourd'hui qualifiées par le pouvoir de « légitimes », après avoir été d'abord minorées, puis méprisées et souvent caricaturées.

Monsieur le ministre, la violence de la politique du président Macron et celle de votre gouvernement, avec des mesures fiscales en faveur des détenteurs de capitaux couplées à des baisses d'aides ou à des augmentations de taxes pour les plus fragiles, ont déclenché cette réaction éruptive. Vous ne pourrez pas dire que le Sénat ne vous avait pas régulièrement mis en garde contre vos excès La réalité est que votre « fabuleuse » théorie initiale du ruissellement ne fonctionne évidemment pas. Le projet de loi de finances que vous nous soumettez aujourd'hui, tout comme d'ailleurs celui de l'année dernière, ne répond pas aux attentes et aux besoins d'une majorité de Français. Il aura malheureusement fallu attendre des émeutes urbaines, par ailleurs insupportables, pour que le Gouvernement, suivant en cela la voie tracée par notre Haute Assemblée, supprime l'augmentation des taxes sur le carburant et reparle, après l'avoir ici méprisée, d'une TICPE flottante.

Encore un effort et vous rétablirez l'ISF, ou tout autre impôt sur le patrimoine : nous ne sommes pas fétichistes. Quoi que vous en disiez, vous ne pouviez pas vous priver, ne fût-ce que moralement, de cette recette tant que nos comptes publics n'étaient pas rétablis et que vous demandiez des efforts à l'ensemble de la Nation. Par charité, je ne m'appesantirai pas sur la demande de suppression de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, une demande par la majorité sénatoriale, mais curieusement et discrètement remisée cette année. J'en viens au texte que nous votons ce jour, c'est-à-dire le texte largement amendé par la majorité sénatoriale. Cela ne surprendra personne au sein de cet hémicycle, nous considérons que le résultat du travail parlementaire conduit par la majorité sénatoriale ne permet pas de répondre aux questions qui nous sont posées aujourd'hui. Chers collègues de la majorité sénatoriale, il faudra qu'un jour vous sortiez enfin de l'ambiguïté dans laquelle vous vous délectez ! Car si le Gouvernement est à l'origine de l'étincelle de ce mouvement social, la gauche comme la droite républicaine doivent clairement expliciter leurs positions.

demander, en même temps pour le coup, sur chaque mission toujours plus d'économies tout en réclamant plus de services publics et de proximité ? Oui, je vous le dis, mes chers collègues, il vous faut maintenant sortir des postures pour afficher une politique d'ensemble claire et crédible ! Imposture ! Pour notre part, durant l'examen de ce projet de loi de finances, nous avons systématiquement gagé nos propositions de dépenses nouvelles. Nous vous avons de nouveau suggéré la réintroduction de l'ISF, appelée de ses voeux par la grande majorité des Français, que vous ne voulez pas entendre, et la suppression de la. Non seulement vous vous y refusez, mais vous trouvez de plus le moyen, avec la complicité de la majorité sénatoriale- il faut le dire -, de diminuer encore l'effet de l'. Nous vous avons aussi suggéré de ne pas transformer le CICE en baisse de charges, et de récupérer ainsi 20 milliards d'euros. Cette mesure risque d'ailleurs d'être utile aujourd'hui pour rééquilibrer vos comptes 2019. Car nous serons vigilants pour que l'on n'assiste pas à un bonneteau fiscal. Les Français ont déjà pu avoir l'impression que la baisse de taxe d'habitation pour la classe moyenne

Pour notre part, nous le souhaitons, et nous y participerons. Nul doute que les Français l'attendent. Au Gouvernement de mieux associer et écouter le Parlement. Vous auriez, monsieur le ministre, beaucoup à mes chers collègues, vous voterez tout à l'heure un budget qui connaîtra dans les jours à venir des modifications majeures. Rendez-vous donc pour la deuxième lecture. Le groupe socialiste et républicain votera sans surprise contre ce projet de loi de finances pour 2019. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, personne, dans cet hémicycle et au-delà, ne se félicitera des conditions dans lesquelles le Sénat a dû cette année examiner le budget de la République. Je ne reviendrai pas sur un malheureux qui a trop pesé sur l'entame de nos discussions. Nous nous sommes déjà exprimés sur ce point, et nos débats ont d'abord besoin de dignité. Bravo ! Ce qui importe surtout, bien au-dessus de ces basses billevesées, c'est de répondre à la crise politique, sociale et sociétale que nous vivons. C'est d'écouter avec la plus grande attention la souffrance exprimée par beaucoup de nos compatriotes, leur volonté de vivre dignement de leur travail. C'est d'apporter des solutions pratiques aux préoccupations qui émergent. C'est, au final, de donner tout leur sens à notre mandat d'élus de la République et aux responsabilités qui en découlent. Oui, il y a bien urgence à apporter des réponses claires et concrètes à ce que beaucoup de nos concitoyens vivent comme une profonde injustice économique et sociale Nous y voyons la conséquence de politiques publiques déconnectées des réalités du quotidien depuis trop longtemps, de décisions incompréhensibles du citoyen, sédimentées dans la plus pure logique technocratique. Ce n'est pourtant pas faute, pour notre groupe, de s'être battu depuis des années en faveur d'une véritable réduction des inégalités, à commencer par celles qui fracturent nos territoires. Je pense ici à l'hyper-ruralité, chère à notre collègue Alain Bertrand. La hausse de la fiscalité des carburants, que le Sénat n'a heureusement pas votée- comme quoi, il a toute son utilité dans notre démocratie ! -, n'en est que le dernier symbole.

et celle qui a peur du chômage, du déclassement social, qui se sent oubliée, pour ne pas dire méprisée, par les gouvernants, dont la porosité avec la haute fonction publique est délétère Les Français qui s'expriment aujourd'hui par la violence nous avaient pourtant lancé des avertissements que bien peu ont entendus par leur vote contestataire, puis par leur abstention et, désormais, par des actes que nous devons interpréter comme une défiance profonde à l'égard de tout ce qui ressemble à une institution. Mes chers collègues, chacun peut porter un jugement détaillé sur le train de mesures annoncé hier soir par le Président de la République. Elles sont désormais dans le champ du débat démocratique. Nous n'avons d'ailleurs pas perdu de temps en débattant tout à l'heure de la prime d'activité. D'autres discussions arriveront très vite. Le groupe du RDSE va se prononcer au vu de tous ces éléments. Bien entendu, nous avons obtenu le vote d'un certain nombre de nos propositions, parmi lesquelles la suppression de l'abattement des journalistes les mieux payés, c'est-à-dire ceux qui touchent plus de 6 000 euros par mois, la redevance des concessions hydroélectriques,

Mais la grande majorité d'entre nous ne pourra pas approuver une loi de finances amputée des crédits de sept missions. De plus, le budget dont nous discutons est obsolète avant même son vote, étant donné les annonces du Président de la République. C'est pourquoi la très grande majorité de mon groupe s'abstiendra, quand quelques-uns s'opposeront au texte, et un le votera. C'est cela, la liberté de vote au sein ! Je sais que certains ici nous l'envient secrètement ! Nous ne pouvons pas non plus poursuivre nos débats sans souligner que le vote d'un budget est au fondement de notre démocratie représentative. Historiquement et philosophiquement, c'est bien par l'acceptation de la levée de l'impôt qu'est née la notion même de Parlement. Or le consentement à l'impôt est aujourd'hui malmené, voire remis en cause, par certains de nos concitoyens, au point de violemment mettre sous tension notre unité nationale. Mon groupe, qui revendique fièrement l'héritage de Georges Clemenceau et de Joseph Caillaux, ne peut évidemment accepter de telles dérives. Nous subissons aujourd'hui les effets de décennies de technicité, d'opacité, de mitage fiscal par la multiplication des niches, au point de rendre notre système incompréhensible, donc inacceptable. Le signal que nous adressent nos compatriotes est aussi qu'il n'est plus possible de continuer dans cette impasse. Revenons donc à la signification profonde de l'impôt, celle de l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : une « une « contribution commune [ ...] également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Redonnons de la lisibilité et de la simplicité à notre édifice fiscal, de telle sorte que nos concitoyens comprennent les efforts qui leur sont demandés et prennent conscience qu'ils participent collectivement à la vie de la Nation. Arrêtons avec une fiscalité vécue comme punitive et socialement injuste ! L'impôt doit redevenir l'outil de citoyenneté qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Il est temps que ceux qui concourent à l'élaboration de l'action publique en prennent la mesure, afin que notre démocratie s'adapte, à la vitesse qui est la sienne, aux évolutions de notre société, reste à l'écoute des Français et essaye de les réconcilier avec l'impôt ! Le Sénat

Sénat a adopté. La parole est à M. le président de la commission. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'heure où nous achevons nos travaux sur le projet de loi de finances pour 2019, je voulais rappeler combien notre assemblée s'est mobilisée pour l'examen de ce texte. Nous y avons consacré 120 heures de séance publique et 216 heures de réunion en commission des finances et en auditions préparatoires des rapporteurs spéciaux. Nous aurons examiné 2 029 amendements, contre seulement 1 363 Le calendrier budgétaire a pu être tenu, malgré les nombreuses vicissitudes qui ont marqué l'examen du texte : le report de certaines discussions de missions budgétaires le week-end en conséquence de votre malheureux, monsieur le ministre de l'action et des comptes publics, l'insertion d'un débat- nécessaire -sur la fiscalité écologique et le pouvoir d'achat avec le Premier ministre au milieu de l'examen des missions budgétaires et, hier encore, les annonces du Président de la République, qui bouleversent une nouvelle fois les équilibres du budget. s'ajouter les effets de l'absence de collectif de fin d'année, qui expliquent en partie « l'inflation » de taille de ce projet de loi de finances. Gageons cependant que nous aurons très prochainement à nous retrouver pour examiner un nouveau collectif budgétaire, tant l'examen du projet de loi de finances pour 2019 présenté par le Gouvernement aura mis en lumière

Je n'oublie pas l'ensemble de notre administration, les services de la commission des finances et des commissions saisies pour avis, ainsi que nos collaborateurs et les professionnels de nos groupes politiques.

La séance est reprise. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution visant à préserver l'ordonnancement juridique relatif au port du voile intégral dans l'espace public présentée, en application de l'article 34-1 de la Constitution, par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues

l'actualité n'épuise pas tous les sujets. Si nous avons tenu à déposer cette proposition de résolution, c'est tout simplement parce que nous pensons que, parfois, il faut réagir. On ne peut pas se taire, On ne peut pas se taire, on ne peut pas faire comme si on n'avait rien vu ni rien su. On ne peut pas se taire non plus comme si on devait seulement opposer le silence à ce qui est de l'ordre de l'inacceptable. De quoi s'agit-il ? Après la plainte de deux femmes

Ce grillage en tissu efface, retranche et diminue. Il efface parce qu'il fait disparaître l'identité et l'individualité des femmes. Il les efface de l'espace public. Il les retranche ensuite

la femme en image incarnée du refus de la figure, alors même que l'islam refuse toute notion d'image ! Enfin, non seulement il efface, non seulement il retranche, mais surtout il diminue la femme en

la valeur de l'égalité de l'homme et de la femme, c'est-à-dire la valeur de la dignité humaine. Elle s'oppose aussi à la valeur de l'universalité de la loi, cette valeur qui fait que nous avons, en France, une communauté civique, une amitié civique. Dans notre pays, la fraternité n'est pas une fraternité d'ordre religieux, c'est une fraternité civique. Aucune de nos communautés, religieuses ou autres, ne saurait s'inscrire à l'intérieur d'un cercle de feu pour se retrancher

de dénoncer le cadre idéologique dans lequel s'enferment un certain nombre d'institutions internationales. Ces institutions internationales, et c'est le cas du Comité des droits de l'homme des Nations unies, se servent de la rhétorique des droits de l'homme pour développer une conception radicale de l'individualisme et du multiculturalisme. Au nom, en réalité, d'une sorte d'exaltation libérale libertaire de la liberté,

du droit est très différente de notre tradition républicaine. Elle atteint à la fois le concept de laïcité puisqu'elle place très haut les droits des individus, au-dessus de tout

lui-même. Je le cite fidèlement : « Même si cette constatation n'a pas, en droit, de force contraignante, l'autorité qui s'y attache de fait constitue un facteur nouveau de déstabilisation de la jurisprudence. Il poursuit : « En réalité, ce phénomène d'internationalisation appelle la culture judiciaire et juridique française à entrer en synthèse avec la culture anglo-saxonne.

c'est une zone grise, un droit jurisprudentiel, qui s'oppose, en réalité, à la démocratie nationale. Très bien ! On le voit en France avec la crise des « gilets jaunes », mais aussi en Europe, au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre avec le Brexit. Ces crises, ces insurrections électorales

nos valeurs et notre attachement aux libertés individuelles, notamment celles des femmes. Ajoutons à cela quarante années de couardise et de compromissions de la classe politique avec les islamistes, et vous obtenez la France des terroirs, des clochers et de Marianne transformée en France terreau de la charia et du voile intégral Ce voile intégral n'est rien d'autre, mes chers collègues, qu'un acte politique posé par des extrémistes islamistes, qui utilisent nos libertés pour mieux les combattre. De la France fille aînée de l'Église à la France petite-fille de l'islamisme, il n'y a qu'un voile ! Pendant que vous palabrez, les barbus agissent. Pourtant, ils ne sont forts que de notre faiblesse. Le port de la burqa est une violence insupportable faite aux femmes, une étape dans la volonté de conquête de l'âme et du corps de notre nation par des fanatiques qui s'engouffrent dans les failles de notre droit pour imposer leur droit, la loi islamique, aidés en cela par des officines internationales d'idéologues qui bafouent les libertés des femmes. De ce constat accablant que chaque Française peut voir et même subir au quotidien, je crains que ce gouvernement n'ait tiré aucune leçon. L'urgence absolue de stopper toute immigration n'est pas à l'ordre du jour, puisque le Président de la République a fait ratifier, en catimini, le pacte mondial sur les migrations de Marrakech, de Marrakech, acte de haute trahison qui achèvera l'entreprise de submersion de notre pays par des millions de migrants, avec, en leur sein, des milliers de fanatiques qui ont la liberté des femmes en détestation. Cessons tout masochisme et déni de la réalité ! Non, monsieur le ministre de l'intérieur, le fichu de nos grands-mères n'a rien à voir avec ce voile qui nie la femme jusqu'à l'enfermer dans un tissu carcéral Ici, ce n'est pas Kaboul, nous sommes en France, à Paris, capitale mondiale de la mode. Ici, les femmes, nous les voulons et nous les aimons en pantalon, en robe, en jupe, en short, en maillot de bain. Nous aimons voir leurs cheveux, nous voulons voir leur visage, leur sourire. Nous les voulons mères au foyer, chefs d'entreprise, saintes héroïnes de la patrie, parlementaires.

domaine des possibles ! Les femmes, ici, nous les voulons et nous les aimons libres ! En ce centième anniversaire de la grande victoire, n'oublions jamais, mes chers collègues, qu'à l'arrière, l'arrière, dans leur foyer mais aussi dans les champs, dans les usines, dans les hôpitaux, ce sont les femmes qui ont porté le pays à bout de bras ! Sans le dévouement des femmes, les hommes au front n'auraient jamais tenu ! Sans les femmes, la France ne serait plus française plus française ! Alors, pour la France, fille aînée aussi de la liberté, ne tergiversons plus ! Ne reculons plus face à l'obscurantisme islamiste ! Redevenons maîtres chez nous : dévoilons une bonne fois pour toutes la République

Le groupe Les Républicains nous invite à débattre de la dissimulation du visage dans l'espace public et de la réaffirmation des dispositifs votés en 2010. Passée la mention d'autres voies et moyens de dissimuler le visage dans l'espace public- la cagoule,

n'a aucune force contraignante dans l'immédiat, mais peut occasionner- je partage sur ce point la position du président Retailleau -des litiges et offrir un terreau favorable à toutes les dérives et victimisations qui peuvent en découler. Répéter une fois de plus les principes républicains du vivre ensemble n'est jamais un rappel de trop. Toutefois, lorsque l'on connaît la force exécutoire des résolutions de l'ONU, je ne crois pas qu'il y ait franchement de grands risques dans l'immédiat, que ce soit pour les constructions illégales dans des territoires occupés

particulier, il serait opportun qu'avant d'engager la France dans des accords aussi importants le Gouvernement consulte le Parlement. Eh oui ! Cette remarque est aussi valable pour les conventions fiscales.

Les Républicains et l'ensemble de la représentation sénatoriale, une mission d'information sur l'islam. La démarche et la volonté de la France s'inscrivent dans un mouvement international convergent, qui s'oppose

Aux Émirats arabes unis, pour d'évidentes raisons de sécurité qui ont présidé au vote du texte de 2010, il est absolument interdit aux femmes travaillant dans certaines administrations de se couvrir le visage ; c'est le cas dans les aéroports, les centres stratégiques, etc. Au Koweït, les femmes qui portent le niqab n'ont tout simplement pas le droit de conduire, ce qui paraît logique. Plus près de nous, le Maroc et la Tunisie ont non seulement interdit le port du niqab, mais aussi sa fabrication.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public concerne non pas quelques centaines ou quelques milliers de personnes, de façon anecdotique, mais notre société tout entière et l'idée que l'on peut se faire de la France. Cette loi est d'autant plus fondée que les autorités religieuses musulmanes, au plus haut niveau, ne rangent pas le port du voile intégral parmi les prescriptions de l'islam, ce qui atteste que cette loi est dirigée non pas contre une religion, mais contre des dérives fondamentalistes, ce qui est totalement différent. En mettant en cause la relation à autrui et la réciprocité d'un échange, la dissimulation du visage dans l'espace public s'oppose directement aux exigences du « savoir vivre ensemble », exigences qui s'imposent à chacun, quelle que soit sa confession. Oui, l'échange social implique d'apparaître à visage découvert dans l'espace public, quand la dissimulation paraît contraire au principe de fraternité et, au-delà, au principe de civilité. Elle marque le refus d'entrer en relation avec autrui ou, plus exactement, d'accepter la réciprocité et l'échange, puisque cette dissimulation permet de voir sans être vu. De plus, au-delà de la mise en cause de la relation à autrui, la dissimulation du visage porte directement atteinte à la dignité de la personne, ce qui constitue une base constitutionnelle incontestable pour l'interdiction prévue, d'autant qu'elle est limitée à l'espace public. De même, le Conseil d'État a relevé que le respect de la dignité de la personne humaine fait partie intégrante de l'ordre public. Le 27 juin 2008, il avait ainsi rejeté la requête d'une Marocaine qui s'était vu refuser l'accès à la nationalité française en raison de sa pratique religieuse radicale, incluait le port de la burqa. L'ordre public est également mis en cause du fait de l'impossibilité d'une identification, qui concerne d'ailleurs tous les modes possibles de dissimulation du visage et toutes les justifications, alors même que les préoccupations de sécurité sont maximales pour nos concitoyens. Ainsi, en 2010, un choix de société a été fait. Aujourd'hui il paraît impérieusement nécessaire de le préserver et de le réaffirmer avec force, dans la mesure où celui-ci semble être menacé. En effet, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a adopté, le 22 octobre 2018, des « constatations », à la suite de la plainte de deux femmes verbalisées en France pour leur port du voile intégral sur la voie publique. Celui-ci a estimé que la loi de 2010 portait atteinte « au droit des deux plaignantes de librement manifester leur religion » et qu'elle constituait, dès lors, une discrimination à caractère religieux. Comme l'indiquent les auteurs de la proposition de résolution, « cette interprétation de la protection des droits de l'homme aboutit de fait à favoriser la négation des droits des femmes et remet frontalement en cause notre conception de leur place dans la société

de façon très claire : « Les autorités nationales jouissent d'une légitimité démocratique directe et [ ...] se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, même prétendument volontaire ou accepté, le port du voile intégral ne consiste en vérité qu'en une forme de réclusion publique. Il n'existe aucune liberté dans le fait de dissimuler son visage. La dignité est l'une des premières libertés dans la patrie des droits de l'homme ; c'est notre héritage humaniste. Aussi, à l'heure où les Français s'interrogent sur le devenir de la Nation et sur l'avenir de ce qu'ils sont, il est de notre responsabilité de faire preuve d'une extrême vigilance et de réaffirmer les valeurs que nous avons en partage et qui sont le fondement de notre volonté de construire un destin commun. Notre devoir est de parler d'une seule voix pour manifester notre attachement unanime à la République, à ses principes et à ses valeurs. En tant que parlementaires, il nous revient aussi de garantir la pérennité de nos valeurs, lesquelles façonnent un modèle qui a fait notre pays et qui fait aussi son image, un modèle qui fonde notre pacte social et forge notre identité. Il nous revient d'être dignes des exigences attachées à l'honneur d'être Français et au privilège de vivre en France.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la question du port du voile dans les lieux publics ne date pas d'aujourd'hui. En 2003, déjà, la commission Stasi l'examinait et concluait ainsi ses travaux : « Dans la conception française, la laïcité n'est pas un simple " garde-frontière " qui se limiterait à faire respecter la séparation entre l'État et les cultes, entre la politique et la sphère spirituelle ou religieuse. L'État permet la consolidation des valeurs communes qui fondent le lien social dans notre pays. » Des pressions s'exercent sur des jeunes filles pour les contraindre à porter un signe religieux, parfois pour les enfermer dans un vêtement. La République ne peut rester sourde à leurs cris de détresse. Aujourd'hui, Aujourd'hui, la question est non plus la liberté de conscience, mais l'ordre public. La montée inexorable du communautarisme et de l'intégrisme dans les quartiers les plus fragiles de notre République, que j'ai pu constater quand j'étais ministre de la ville, a conduit en 2010 les parlementaires- on l'a dit -à voter une loi interdisant le port du voile intégral sur la voie publique. Dans une lettre de mission, le Premier ministre demandait au Conseil d'État d'étudier des solutions juridiques permettant de parvenir à une interdiction du port du voile intégral qui soit la plus large et la plus effective possible, tout en rappelant, bien sûr, la nécessité de ne pas blesser nos compatriotes de confession musulmane.

par vos fonctions antérieures et présentes -pour savoir que la menace terroriste n'a jamais été aussi présente sur notre territoire. Nous avons évité bien des attentats, grâce au courage des services de la République que vous avez, pour partie, La société française et ses représentants pensent que le voile intégral n'a rien à faire sur la voie publique, d'abord pour une raison d'ordre public- Bruno Retailleau l'a dit -, ensuite et surtout au nom de la dignité de la femme. Ce comité Théodule des droits de l'homme des Nations unies, en estimant que la loi interdisant la dissimulation du visage est une atteinte à la liberté religieuse, fait un contresens total. Il méconnaît civils et politiques du 16 décembre 1966, qui prend en compte les spécificités des sociétés des pays signataires et précise que la liberté de religion peut être limitée dans un but de protection de l'ordre public, de la sécurité ou de la santé publique. Le port du voile intégral n'est pas acceptable dans le pays des droits de l'homme, qui est aussi, on l'a dit, celui des droits de la femme. Par la soumission de la femme qu'elle manifeste, cette pratique est contraire aux principes fondamentaux de notre identité nationale, au premier rang desquels l'égale dignité de l'homme et de la femme et l'existence d'un espace public de dialogue. L'idée qu'il puisse exister un vêtement du visage correspond à une conception des rapports humains qui n'est absolument pas tolérable sur notre sol. Cela reviendrait à considérer que les femmes ne sont pas dignes d'être vues ou d'entrer en relation avec les autres, au même titre que les hommes. Laisser se développer une telle pratique conduirait à favoriser l'amalgame entre la religion musulmane et l'islamisme intégriste. On a d'ailleurs souligné à plusieurs reprises que plusieurs représentants de la religion musulmane avaient toujours été très clairs sur ce sujet. Revenir sur cette législation après les crimes commis par Al-Qaïda, par Boko Haram ou par Daech, après le génocide et les viols commis sur les populations azéries, après l'attentat du Bataclan serait une insulte adressée à toutes les familles des victimes. Monsieur le secrétaire d'État, dans ma commune de 30 000 habitants, un jeune homme de 29 ans a été assassiné au Bataclan. Je connaissais très bien ses parents, et je suis allé moi-même leur annoncer sa mort. Ils ne comprendraient en aucun cas que l'on puisse revenir sur une telle législation. Revenir sur cette législation après de telles provocations, ce serait adresser à la nation française un message de tolérance face à l'intolérable. Revenir sur cette législation, ce serait envoyer un signal profondément désespérant aux millions de femmes qui espèrent leur émancipation partout dans le monde. Ce serait pour la France déchoir de son rôle de défenseur des droits fondamentaux. C'est toute la République qui dit non au voile intégral. Voilà pourquoi nous soutenons pleinement la proposition de résolution de notre président Bruno Retailleau, et nous appelons, bien sûr, le Gouvernement

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il y a bien longtemps que le port du voile intégral ne s'était pas invité dans le débat politique. Avec cette proposition de résolution, il y refait son apparition. Examinons les faits. La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public fut adoptée à la quasi-unanimité par les deux chambres. Le Conseil constitutionnel la jugea conforme à nos principes, en particulier à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. De même, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, déclara que cette loi respectait

saisi par deux plaignantes, estime que cette loi de 2010 porte atteinte « au droit des deux plaignantes de librement manifester leur religion ».

Certes, dans le passé, ce comité s'était prononcé sur l'aspect discriminatoire des règles de neutralité religieuse dans la fameuse affaire de la crèche Baby Loup. Cet avis avait trouvé un écho au niveau juridictionnel, le premier président de la Cour de cassation, comme vous l'avez rappelé, monsieur Retailleau, ayant prévenu que l'institution qu'il dirigeait tiendrait compte de cette interprétation en raison de l'autorité qui s'y attachait de fait. Cette position est finalement assez constante et les juges s'appuient volontiers sur des avis non contraignants pour interpréter la loi. Sauf que, dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas de l'espace public. Bref, ce magistrat aurait pu prendre une autre décision. La loi est là, elle est issue d'une volonté démocratique forte établie par les représentants du peuple, la branche législative du pouvoir. La CEDH avait reconnu et réaffirmé : « Il apparaît ainsi que la question de l'acceptation ou non du port du voile intégral dans l'espace public constitue un choix de société. » La jurisprudence n'est pas modifiée par la décision du Comité des droits de l'homme, l'ordonnancement juridique est intact, et la volonté de la société d'établir une règle du vivre ensemble dans l'espace public préservée. Enfin, limiter nommément cette question d'application de la loi au seul voile islamique, alors que la loi du 11 octobre 2010 a permis d'affirmer et de sanctuariser le principe fondamental selon lequel « la République avance à visage découvert », me paraît constituer, mes chers collègues, une tentative de soulever un débat qui ne devrait plus avoir lieu d'être, à des fins qui risqueraient de s'éloigner de la préoccupation juridique pour glisser vers une intervention plus politique. Pourquoi pas ? Puisque vous voulez parler du voile, parlons-en Le port du voile intégral est-il un mode d'expression d'une foi religieuse, à savoir l'islam, ou bien une simple tradition vestimentaire imposée, dans certaines terres d'islam, aux femmes contre leur gré, parfois même sous peine de mort ? En tout cas, si le Coran lui-même recommande une certaine pudeur vestimentaire pour les femmes, comme d'ailleurs pour les hommes, je n'y ai jamais lu une quelconque obligation du voile intégral ; il ne contient même pas le mot « ». Il n'y a d'ailleurs dans le Coran que quatre versets sur ce sujet. La seule partie du corps féminin qu'il est recommandé de couvrir est la poitrine. Selon Asma Barlas, universitaire américaine d'origine pakistanaise, le port d'un voile intégral qui couvre le visage « est absolument contraire à l'esprit du Coran ». Elle poursuit : « J'en veux pour preuve que les femmes doivent accomplir le hadj, le pèlerinage rituel, à visage découvert. Selon Mme Barlas, la question du voile cristallise d'autres craintes ; si les femmes sont opprimées dans le monde islamique, c'est le fait des hommes, pas de la religion. C'est bien là qu'est le problème de fond. L'islam n'impose pas le voile intégral. Ce dernier est devenu une marque identitaire, voire une provocation face à notre tolérance occidentale issue de la philosophie des Lumières. Si c'est cela le retour du spirituel annoncé par Malraux ... Permettez-moi de n'y voir qu'obscurantisme, rabaissement de la femme et intolérance ! Ce n'est pas comme cela que je vois l'islam de France et, au-delà, l'islam tout court. Ce n'est pas parce que certains pays musulmans ont inventé le voile intégral, qu'on l'appelle burqa ou niqab suivant le « modèle »- passez-moi l'expression -et surtout le pays, que nous devons l'accepter dans notre pays laïc, lequel tolère, ,aussi le multiculturalisme, même si le mot peut avoir une consonance pour certains. Restons ouverts à cette grande religion qu'est l'islam en lisant ou relisant le Coran avec le regretté Mohammed Arkoun, grande figure de l'islamologie contemporaine, ou en pensant le politique avec Abdou Filali-Ansary, directeur de l'Institut pour l'étude des civilisations musulmanes de Londres, qui réfute jusqu'à l'idée même d'un État islamique. Soyons intraitables face à des dérives radicales, voire fanatiques, et de toute façon humiliantes pour les femmes. Disons-le, la présence dans l'espace public de femmes intégralement voilées a heurté la vision qu'avait notre pays de la place des femmes en son sein

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la laïcité française, dans ses principes et ses modalités d'application, demeure une spécificité de notre République et ses conceptions originales doivent être collectivement défendues, sur notre sol et dans les instances internationales. La Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe n'ont jamais, dans leurs nombreuses décisions, contesté les législations ou les décisions judiciaires fondées sur de tels préceptes. En revanche, le Comité du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a parfois manifesté de l'incompréhension ou de l'opposition à l'égard de la laïcité française. Cette proposition de résolution aurait pu être l'occasion de lui rappeler notre attachement collectif à cet élément fondamental de notre socle républicain, d'en défendre les principes et d'en promouvoir la valeur universaliste. Nous regrettons donc vivement que le mot « laïcité » n'y soit jamais cité, ni dans l'exposé des motifs ni dans le texte même. À propos des constatations du Comité des droits de l'homme des Nations unies publiées le 22 octobre 2018, il convient, en préambule, de préciser qu'elles n'ont aucune conséquence juridique sur le droit français. En aucune façon, elles ne modifient l'ordonnancement juridique national ou n'atténuent la portée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Les mesures proposées aux alinéas 14 et 15 de la présente proposition de résolution sont donc sans objet. Néanmoins, je pense qu'il aurait été utile pour nos débats de reprendre ici certaines des observations présentées par la majorité des membres de ce comité. En effet, plusieurs d'entre eux partagent l'idée que le voile dissimulant totalement le visage, appelé niqab, est « discriminatoire ». Ils estiment que « le port du voile intégral est une pratique traditionnelle par laquelle les hommes ont asservi les femmes sous couvert de préserver leur " pudeur les empêchant ainsi d'occuper l'espace public au même titre que les hommes ». De même, le Comité, dans sa décision, reconnaît à l'État français le droit de « promouvoir la sociabilité et le respect mutuel entre les individus, dans toute leur diversité, sur son territoire, et conçoit que la dissimulation du visage puisse être perçue comme un obstacle potentiel à cette interaction »., ce qui est contesté par ce comité, c'est moins la mesure elle-même, l'interdiction du voile intégral, que la disproportion de la restriction de circulation, par rapport à un objectif qu'il estime mal défini par la loi. Sur ce dernier point, la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public aurait pu, il est vrai, être plus explicite. Son premier article dispose : « Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». En revanche, l'exposé des motifs est beaucoup plus précis puisqu'il considère, avec justesse, que « la dissimulation du visage dans l'espace public est porteuse d'une violence symbolique et déshumanisante, qui heurte le corps social » et que le voile revient « à nier l'appartenance à la société des personnes » qui le portent. Fondamentalement, l'objet même de la loi est non pas la nature du bout de tissu porté par un individu, mais la position politique qui dénie à une femme ses droits de citoyenne, conformément à des traditions religieuses qui s'imposeraient à l'ordre républicain. Il s'agit non pas de réglementer la dissimulation du visage, qui pourrait concerner, de la même façon, la femme intégralement voilée et l'individu qui souhaiterait cacher son identité aux forces de sécurité, mais de réaffirmer, dans l'exercice de la citoyenneté à laquelle nul ne peut renoncer, la primauté des lois de la République sur les croyances ou les systèmes de pensée qui lui sont extérieurs. Là est bien l'essence de la laïcité. À ce propos, j'aimerais rendre hommage au courage de M. Yadh Ben Achour, juriste tunisien et membre du Comité aux droits de l'homme, qui a souhaité exprimer avec force son opposition à la décision de cette instance. C'est vrai ! Ses arguments ont été repris en annexe de la décision et méritent d'être cités de nouveau Je le cite Or, en soi, le niqab est un symbole de stigmatisation et d'infériorisation des femmes, par conséquent contraire à l'ordre républicain [ ...]. Les défenseurs du niqab enferment la femme dans son statut biologique primaire de femelle, objet sexuel, chair sans esprit ni raison, responsable potentiel du désordre cosmique et du désordre moral, et qui doit donc se rendre invisible au regard masculin et être pour cela quasiment interdite de l'espace public. Un État démocratique ne peut permettre une telle stigmatisation [ ...]. » M. Yadh Ben Achour, en tant que Tunisien et professeur de droit public, observe que les droits de l'homme se heurtent à « l'arc référentiel » de la croyance islamique, selon laquelle l'ordre du monde ici-bas est comme subordonné à celui de l'au-delà et que les droits de Dieu sont supérieurs à ceux des individus. Pour lui, la religion ne peut être autoréférentielle. Elle doit se soumettre à la raison universelle. Alors que nous allons peut-être débattre prochainement des lois de bioéthique, notre assemblée est-elle prête à reconnaître entièrement cette soumission ? Êtes-vous prêts, chers collègues, à considérer que la laïcité est la condition première de l'émancipation des femmes et de l'affirmation de leur liberté à disposer librement de leur corps, y compris lors de la procréation ? La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, notre République est laïque.

Comme notre République est laïque, elle garantit à chacune et à chacun le droit d'exercer, de vivre sa religion, le droit de dire et de manifester ses opinions et ses convictions. Comme notre République est laïque, les religions doivent être exercées par chacune et chacun dans le respect de la loi. La loi républicaine s'impose à tous parce que, laïque, elle permet à chacune et à chacun d'exercer librement sa religion, de faire vivre et d'exprimer ses convictions.

Il est bavard, monsieur Karoutchi, il n'est pas le seul d'ailleurs ... Ce comité n'a aucun pouvoir : il ne prend pas de décisions, il fait des constatations- c'est le terme juridique.

Je partage beaucoup de ce qui a été dit par MM. Amiel et Ouzoulias. Notre groupe, après en avoir délibéré, ne prendra pas part au vote, et je tiens à expliquer pourquoi. pourquoi. Bien entendu, nous sommes totalement opposés au port de la burqa ; nous sommes cent fois, mille fois, partisans de la loi de 2010, que nous avons votée et que nous pensons absolument nécessaire. Simplement, est-il utile, en cette occasion, de revenir sur quantité de sujets le communautarisme, le statut des femmes, l'intégrisme, le terrorisme et nos valeurs culturelles ? Oui ! On peut le faire, bien sûr, et nous partageons beaucoup de choses à cet égard. Néanmoins, très concrètement,

va donner suite aux constatations de ce comité qui n'a aucun pouvoir. Personne ne le pense. Et s'il advenait dans notre pays qu'un gouvernement ait cette idée, tous les groupes du Parlement se dresseraient, du moins je l'espère,

c'est que l'interdiction de couvrir intégralement le visage repose sur deux principes, et deux principes seulement, ce en quoi elle a une valeur universelle.

que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme doivent primer sur ce comité qui n'a aucun pouvoir. Cela me paraît aller

de 2010 : c'est une loi qui protège les femmes, qui protège l'espace public et qui aide à faire de la société française une société plus pacifiée et plus respectueuse de chacun ; bien sûr, toute personne est libre de porter dans l'espace public un vêtement destiné à manifester une conviction religieuse ; toutefois, la loi peut interdire la dissimulation du visage, dans la mesure où cela est jugé incompatible avec les principes de sécurité et de fraternité qui fondent la société démocratique dans laquelle nous vivons. Tout est dit, mes chers collègues, et nous devons remercier la Cour européenne des droits de l'homme d'avoir pris une si forte décision. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 25 octobre dernier, lorsque j'avais interrogé Mme la garde des sceaux sur l'avis du Comité des droits de l'homme de l'ONU relatif à la loi de 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, je réagissais fortement aux commentaires de la presse qui ne s'était pas documentée sur la portée de cet avis ... Cela arrive ! ... et à quelques propos du premier président de la Cour de cassation, que Bruno Retailleau a cités. Si les membres de mon groupe et moi-même ne nous étonnons guère des constatations hostiles d'un comité composé de 18 experts internationaux, ... Experts ... ... il est en revanche plus inquiétant que la plus haute juridiction française instille quelques doutes sur la nature de sa mission, en prêtant à ce comité de l'importance. Faut-il rappeler que, conformément à l'article 5 du code civil, les juges français ont l'obligation d'être « la bouche de la loi » ? La fin du légicentrisme fait peser sur la loi une présomption de faillibilité qui n'est pas sécurisante pour les citoyens, surtout quand celle-ci a pour objet de garantir un modèle de vie un modèle de vie en société largement partagé, de prévenir les atteintes à l'ordre public ou les inégalités entre les sexes, comme c'est le cas s'agissant de la laïcité. Pour autant, il n'est pas fondé de considérer que le législateur n'a pas pris la mesure des risques de conflits de normes entre les blocs de légalité, de constitutionnalité et de conventionnalité. Il me semble que la mission d'intégration des directives croissantes d'origines diverses à l'État de droit est précisément la prérogative du Parlement, qui l'exerce tous les jours, sur ces travées. À qui revient-il de dire lesquelles de ces influences incarnent l'intérêt général, si ce n'est aux membres du Parlement ? Nos débats se font régulièrement l'écho de telle ou telle jurisprudence pour éviter des incompatibilités inutiles, mais il arrive également que les conflits de normes découlent pertinemment de conflits politiques ou de l'affrontement de différents modèles de pensée. Ce pourrait être le cas du principe de laïcité, si la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, ou une autre instance dotée d'un pouvoir contraignant avait décidé de remettre en cause notre régime de séparation des Églises et de l'État. Ce n'est heureusement pas le cas Sans parler des théocraties, certains modèles concurrents au modèle français cherchent à étendre leur influence dans le monde. Je pense en particulier au modèle anglo-saxon, qui consacre la liberté absolue d'affirmer son identité religieuse, sans en favoriser aucune, comme il reconnaît un pouvoir important aux « communautés ». Selon cette interprétation, l'espace public peut être le lieu de toutes les manifestations religieuses, en particulier vestimentaires. C'est ce modèle que semble vouloir imposer, aujourd'hui, le Comité des droits de l'homme à l'ensemble des États-nations, sans garantie d'ailleurs que sa jurisprudence reste stable, au gré des nominations et recompositions. en émettant un avis contraire aux jurisprudences de la Cour de cassation et de la CEDH, il nuit à l'unité républicaine et menace notre cohésion sociale, déjà mise à rude épreuve. De surcroît, ses avis, ne trouvant pas à s'appliquer devant nos tribunaux, contribuent à nourrir un sentiment d'injustice sans fondement. La proposition de résolution de M. Retailleau et de ses collègues rappelle, avec justesse, que le Parlement était souverain lorsqu'il a adopté, à la quasi-unanimité, la loi de 2010 sur l'interdiction de dissimulation du visage dans l'espace public. Aucune juridiction française ne peut éluder cette réalité, sous l'effet d'une injonction externe non contraignante. Partant de ce même constat, j'incite fortement le Gouvernement à répondre à l'avis du Comité des droits de l'homme, en défendant avec fermeté la pertinence de notre principe de laïcité et l'égalité entre les femmes et les hommes, dans un contexte mondialisé où les individus sont et seront exposés à une plus grande diversité religieuse. Ce principe de laïcité incarne, dans notre modèle républicain, le principe d'égalité, dont découle celui de neutralité de l'État. Ce dernier doit traiter tous les citoyens à égalité de droits, quelle que soit leur religion, dans le respect de la liberté d'expression, de la liberté religieuse, celle de croire ou de ne pas croire, et nous devons, femmes et hommes, pouvoir nous promener où nous voulons, quand nous voulons. De plus, contrairement à ce qu'en disent ses détracteurs, la loi de 1905 reste un cadre satisfaisant pour l'évolution du paysage religieux français et elle n'a été un obstacle au développement d'aucun culte. Les « frottements » constatés ont été des occasions d'affirmer les limites entre « le temps de l'école et le temps de Dieu » et les pratiques religieuses admises ou non dans l'espace public, à l'image de la loi de 2010. Je rappelle que cette dernière a été adoptée par le Parlement pour des raisons de sécurité publique et non pour des raisons de laïcité. J'ai envie de vous poser une question simple, voire simpliste, monsieur le secrétaire d'État : et si nous appliquions les lois ? Les initiatives comme celle du Comité des droits de l'homme de l'ONU fragilisent le principe de laïcité et l'équilibre pacifique séculier dans notre pays. Après la clarification de l'objectif visé par M. Retailleau et ses collègues, le groupe du RDSE votera cette proposition

secrétaire d'État, mes chers collègues, voilà deux mois, je défendais dans cet hémicycle la nécessité de combattre plus efficacement le port du voile intégral, qui heurte nos valeurs les plus fondamentales. N'ayant plus d'argument à opposer à cette interdiction, certains invoquent le Comité des droits de l'homme des Nations unies, qui, par ses observations, a critiqué l'interdiction de la burqa prévue par notre législation. Cette proposition de résolution entend justement remettre les choses à leur place. Je salue l'initiative du président Bruno Retailleau, qui a rappelé la nécessité, pour notre pays, de se défendre à l'encontre d'accusations lancées dans l'arène internationale. Non, la communauté internationale n'a pas condamné la France ! À tous ceux qui se retranchent derrière les Nations unies, je rappelle, comme tant d'autres avant moi ici, que le Comité des droits de l'homme n'est qu'un organe subsidiaire, une espèce de comité Théodule. Il n'a pas la même autorité que l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité. Il est composé de soi-disant experts, non de représentants des États membres des Nations unies, et les observations qu'il émet ne présentent aucun caractère contraignant. Je rappelle justement que la Charte des Nations unies proclame la souveraineté de ses États membres. Dans cette souveraineté, il y a le droit pour chaque État de définir les infractions pénales, le droit de sanctionner les comportements qui choquent la vie en société. Cela n'a jamais été contesté. Le voile intégral porte justement atteinte à la cohésion de notre société. Le législateur français avait le droit de sanctionner ce comportement, même si je souhaite que l'infraction soit érigée en délit, monsieur le secrétaire d'État. On invoque le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui prévoit notamment la liberté de manifester sa religion.

des « restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui ». Justement, le le législateur avait estimé qu'il y avait une atteinte à l'ordre public, mais également à la dignité de la femme. Le voile intégral est bien une atteinte aux droits fondamentaux ! Comme on nous oppose la liberté de religion, autant rappeler l'exégèse des textes invoqués, qui n'empêchent nullement l'interdiction de certains comportements choquants. Le droit international n'interdit donc pas la prohibition du voile intégral. Cette interdiction ne met pas en cause la liberté de conscience ou de culte, car elle touche à l'ordre public et non à des questions de for interne. Ce sont non pas des convictions que l'on refuse, mais des comportements choquants dans l'espace public. Le port du voile intégral n'est pas seulement une attitude religieuse. Au-delà même d'un acte politique, c'est une pure provocation. Il s'agit de narguer les forces de l'ordre et les valeurs de notre société. Ceux qui défendent le port du voile intégral ne font pas autre chose que de tomber dans un piège. Nous n'avons pas besoin d'idiots utiles, comme le disait le camarade Lénine. En outre, d'autres juridictions ont constaté qu'il n'y avait aucune atteinte aux droits et libertés. Je veux citer la Cour européenne des droits de l'homme. Sa jurisprudence, abondante et sourcilleuse, fait autorité en matière de défense des droits de l'homme. Dans le droit international, ses décisions sont scrutées et analysées avec attention. On ne peut pas la soupçonner de partialité à l'égard de la France. Notre pays est parfois passé sous les fourches caudines des juges de Strasbourg. Comme le souligne justement l'exposé des motifs de cette proposition de résolution, la Cour a rappelé la possibilité pour l'État de faire « respecter les exigences minimales de la vie en société ». Cette position, rendue en 2014, a d'ailleurs été confirmée l'année dernière. Puisque l'on cite le droit international relatif aux droits de l'homme, autant le citer intégralement ! Les juges de Strasbourg ou du Palais-Royal, dont personne ne peut nier l'autorité juridique, ont bien confirmé que les libertés publiques n'étaient pas mises en cause par cette loi. Je peine à comprendre ceux qui refusent à tout prix l'interdiction du port du voile intégral. En réalité, ils se font les défenseurs non de la liberté de conscience, mais bien du communautarisme, qui fragilise notre société. Ils sont les complices de l'islam radical que nous devons combattre. Cette proposition de résolution doit être adoptée. J'invite mes collègues à lui donner l'adhésion la plus large. Il faut résister à toutes les déstabilisations, même médiatiques, à l'encontre de la sagesse du législateur français ! La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la France a-t-elle encore son avenir entre ses mains ? Le peuple français est-il encore souverain ? La loi est-elle encore l'expression d'un destin commun ? La réponse à ces questions sera sans doute négative si l'on apporte une modification à l'ordonnancement juridique actuel relatif au port du voile intégral, comme voudrait nous y contraindre, alors qu'il s'agit d'un simple avis, le Comité des droits de l'homme des Nations unies. Mais que nous reproche-t-on ? D'avoir défini un cadre juridique qui serait discriminatoire et contraire à la liberté religieuse ? C'est une folie ! Car c'est ignorer, tout d'abord, que la France est la patrie des droits de l'homme et qu'elle a donné au monde des valeurs universelles qui ont présidé, notamment, à la création de ce même comité. Quelle plus belle preuve de liberté et de tolérance qu'un pays comme le nôtre, qui reconnaît uniquement des citoyens, sans les distinguer selon leur religion, ni leur couleur de peau, leurs origines ou leurs opinions politiques C'est ignorer, aussi, le principe cardinal de laïcité dans notre République, qui prône non pas l'indifférence des religions, mais la neutralité permettant le vivre ensemble. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État en donne une définition très claire : la laïcité accepte tous les cultes et n'en favorise aucun. Certains ne lisent que la première partie du texte ; dès lors, la République devrait accepter un droit absolu à la différence au nom de la liberté, elle aussi absolue, de croyance. C'est la voie du communautarisme et c'est le parti pris des décisions onusiennes qui nous occupent aujourd'hui. D'autres, encore, ne voient que la deuxième partie de la proposition : la République ne reconnaît aucun culte. C'est une laïcité faite de passivité et d'ignorance du fait religieux. Cependant, à force d'ignorer, le pas est rapidement franchi vers le mépris et le rejet des religions. De la même manière, je m'y oppose. C'est également ignorer les droits de la femme de ne pas subir quelque pression ou domination que ce soit pour se sentir libre de ce qu'elle est et de ce qu'elle veut accomplir. C'est ignorer, ensuite, la légitimité du Parlement et des représentants du peuple souverain de prendre les décisions qui s'imposent pour garantir notre coexistence et l'adhésion au pacte national. C'est aussi lancer un message de défiance à l'égard de nos institutions nationales garantes des libertés de chacun, comme le Conseil constitutionnel, qui avait jugé cette loi conforme au bloc de constitutionnalité. Il est d'ailleurs à noter que, depuis l'adoption du texte, plusieurs voisins européens ont fait le même choix. Seraient-ils, eux aussi, de dangereux obscurantistes ? C'est ignorer, enfin, le danger de l'islamisme radical et politique, qui prône le communautarisme là où nous sommes une Nation. Si l'islam a toute sa place en France, le combat contre toute forme d'intégrisme est une absolue priorité à l'aune des terribles attentats que notre pays a connus et qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. À ceux qui veulent diviser la République et affaiblir ce que nous sommes, nous opposons une unité qui passe par le respect de certaines règles, dont celle qui interdit le port du voile intégral dans l'espace public. Ainsi, mes chers collègues, nous n'avons aucune leçon à recevoir d'un comité, composé d'experts qui n'entendent rien ni à nos traditions républicaines ni à notre volonté de combattre toutes les formes de communautarisme. De la même manière, nous n'avons absolument pas à nous justifier pour conserver notre droit à oeuvrer comme nous l'entendons à l'intérêt général au service de tous les Français. C'est pourquoi, vous l'avez compris, je soutiens évidemment avec force cette proposition de résolution du président Retailleau

Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public a été adoptée le 11 octobre 2010 à la suite de vifs débats en France autour du port du voile intégral. tous rappelé, faisait suite à un très large consensus des parlementaires sur tous les bancs, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Ce consensus montre à quel point cette question est, au-delà des enjeux un enjeu de société, qui nécessitait, hier comme aujourd'hui, l'union des parlementaires, de la majorité comme de l'opposition, avec l'appui du Gouvernement. C'est dans cet esprit que je me présente aujourd'hui devant vous, au-delà des logiques partisanes, pour débattre de la proposition de résolution portée par le président Bruno Retailleau, qui vise à réaffirmer la légitimité et la nécessité de cette loi. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la proposition de résolution qui vous est soumise fait suite aux constatations du Comité des droits de l'homme de l'ONU, lequel a estimé que cette loi, à laquelle nous sommes tous attachés ici, constituait, pour les femmes qui portent le voile intégral, une discrimination à caractère religieux et qu'elle portait atteinte au droit de manifester leur religion. Face à ces constatations, vous souhaitez donc, d'une part, réaffirmer votre attachement à la loi de 2010, d'autre part, appeler le Gouvernement à ne pas donner suite à ces constatations. Sur ces deux points, qui forment le coeur de votre proposition de résolution, la position du Gouvernement est claire. claire. Nous partageons pleinement votre attachement à la loi de 2010, que nul ne souhaite remettre en cause et qui est pleinement conforme aux conventions internationales qui nous lient. Sur ce point, nous sommes toutes et tous d'accord. Cependant, le Gouvernement est aussi attaché au respect de ses engagements internationaux. Or, en l'espèce, le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques prévoit que la France réponde aux constatations du Comité des droits de l'homme lorsque celui-ci formule des critiques à son encontre. Le Gouvernement entendra donc y répondre, fermement,

Vous le savez, la loi du 11 octobre 2010, adoptée à la suite de débats politiques approfondis, s'inscrivait dans une logique de préservation de l'ordre public, plus exactement, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel,

qui peut se satisfaire que des personnes se soustraient, par la dissimulation de leur visage, aux interactions sociales qui constituent le liant d'une vie en société ? Peut-on considérer comme conforme à l'égale dignité de chacun, en particulier à l'égalité entre les femmes et les hommes, et les hommes, une telle attitude, quand bien même elle serait revendiquée comme libre par les personnes concernées ? Face à ces interrogations, la position du législateur, celle de l'État, a été sans ambiguïté il fallait marquer la désapprobation de la Nation à l'égard de telles attitudes et condamner de telles pratiques, mais le faire avec le souci de ne stigmatiser aucune religion et de respecter une stricte proportionnalité. Je tiens à le préciser devant vous, car vous entendez encore comme moi les voix qui, à l'époque, s'élevaient contre une prétendue stigmatisation : il s'agit bien d'une loi sur la dissimulation du visage, et non sur la stigmatisation d'une religion,

tels que la Belgique, l'Italie, l'Autriche ou le Danemark, certains de ces pays ayant suivi notre exemple. L'exemple de notre pays, en la matière, c'est également celui d'une réponse proportionnée et, par là même, pleinement conforme au droit. Cette loi a ainsi prévu une sanction adaptée et proportionnée, à savoir une amende ou l'accomplissement d'un stage de citoyenneté pour toute personne dissimulant son visage dans l'espace public. Ce souci de proportionnalité a d'ailleurs été relevé par le Conseil constitutionnel, qui en a conclu été relevé par le Conseil constitutionnel, qui en a conclu que le législateur avait correctement concilié les préoccupations de l'ordre public et de la liberté religieuse. Dans la continuité de ces objectifs- ne pas stigmatiser et apporter une réponse proportionnée de l'État

générale de la dissimulation du visage, afin que chacun et chacune puissent l'anticiper. La circulaire du Premier ministre du 2 mars 2011 appelait plus particulièrement à mettre ce délai de six mois à profit pour faire connaître le texte et informer les personnes concernées. Mais tracer la genèse de cette loi me conduit naturellement à aborder sa réception par les juridictions et organismes internationaux, notamment la Cour européenne des droits de l'homme et, plus récemment, le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Je tiens ici, avant toute chose, à rappeler que, contrairement à ce que vous écrivez dans l'exposé des motifs de la proposition de résolution, on ne peut pas mettre ces deux instances sur le même plan, la première étant l'une de nos juridictions suprêmes, le second, un simple comité d'experts internationaux. Voilà un peu plus d'un an, le 1 novembre 2017, le Président de la République rappelait, à Strasbourg, l'attachement profond de la France aux droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, et à son instrument le plus efficace de mise en oeuvre qu'est la Cour européenne des droits de l'homme. Cet attachement, le Président l'a souligné, implique aussi notre attachement « à la force obligatoire des arrêts de la Cour ». En l'espèce, cette loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public, qu'en a dit la Cour ? Saisie par une requérante, dans son arrêt de 2014, elle a écarté fermement toute violation de la Convention du fait de l'application de la loi de 2010, dont elle a jugé qu'elle ne revêtait pas de caractère discriminatoire et qu'elle ne portait atteinte ni au respect de la vie privée, ni à la liberté de conscience, ni à la liberté d'expression. Aussi, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la préservation de conditions du vivre ensemble était un objectif légitime et que cette loi entrait dans la marge d'appréciation qui revient, fort heureusement, aux États pour définir ce vivre ensemble- le sénateur Pierre Charon Au contraire, le Comité des droits de l'homme de l'ONU, saisi d'une requête individuelle, a rendu le 22 octobre dernier des constatations sur la loi du 11 octobre 2010, dans lesquelles il estime que l'application de cette loi porte atteinte au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion résultant de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à l'interdiction des discriminations prévue par l'article 26 de ce même pacte.

Organe non juridictionnel, le comité ne reconnaît, à la différence de la Cour européenne des droits de l'homme, pas de marge nationale d'appréciation sur les questions concernant la préservation du vivre ensemble. À cet égard, je me permets de souligner que les récentes constatations du Pacte s'inscrivent résolument dans la continuité de ses orientations traditionnelles. Le Comité s'était ainsi déjà prononcé contre l'obligation de poser tête nue sur les photos d'identité en 2013 et contre l'interdiction, résultant de la loi de 2004, du port de signes religieux ostensibles par les élèves de l'école publique. ces constatations ne sont ni une condamnation de l'État ni une injonction au Gouvernement. En somme, elles ne permettent pas de remettre en cause notre droit national. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, j'entends vos inquiétudes et votre souhait d'adopter la proposition de résolution dont nous discutons aujourd'hui. Cependant, comme je viens d'essayer de le démontrer, ces inquiétudes ne sont pas fondées tant la détermination du Gouvernement à préserver et appliquer cette loi et les jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme est intacte. Vos inquiétudes sont d'autant moins fondées que les constatations du Comité des droits de l'homme de l'ONU sont dépourvues de portée contraignante et n'ont donc pas vocation à bouleverser notre paradigme législatif et juridique actuel. proposition de résolution aurait un caractère contre-productif, en ce qu'elle invite le Gouvernement « à ne pas donner suite à ces constatations ». Or, conformément à la Constitution et à nos traditions en pareille situation, et justement parce que nous défendrons toujours notre vision du vivre ensemble, la France entend répondre aux constatations du Comité des droits de l'homme Vous connaissez comme moi ce dicton populaire : « Qui ne dit mot consent. » Eh bien, la France répondra, car elle ne consent pas : là est notre point d'accord. Monsieur